Monsieur le président,

La parole est à M. Jean-Luc Fichet, rapporteur du groupe de travail. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, malgré les mesures mises en oeuvre par les gouvernements successifs au cours des dernières décennies, la route demeure, en France, la première cause de mort violente. Chaque année, environ 3 500 personnes meurent dans un accident de voiture et 75 000 sont blessées, dont 28 000 grièvement. Ce constat préoccupant appelle une politique publique forte de lutte contre l'insécurité routière. La fixation des vitesses maximales autorisées, le port obligatoire de la ceinture et du casque, l'introduction du permis à points, ou encore l'introduction des radars automatiques sont autant de mesures qui ont permis de mieux sécuriser nos routes. Ainsi, entre 1970 et 2010, la baisse du nombre de morts a été significative, puisque l'on est passé de plus de 17 000 personnes tuées à moins de 4 000. Il semblerait toutefois que nous ayons atteint un palier : malgré de nouvelles mesures, les chiffres de l'insécurité routière ne diminuent plus depuis 2013 et sont même en légère augmentation. Pour répondre à cette inversion de tendance, le Premier ministre a annoncé, le 9 janvier dernier, le lancement d'un nouveau plan de lutte contre l'insécurité routière. Composé de dix-huit mesures, ce plan vise à donner une nouvelle impulsion, afin de faire baisser la mortalité sur les routes. L'objectif annoncé est ambitieux : atteindre moins de 2 000 morts sur les routes d'ici à 2020. L'une de ces mesures a focalisé le débat public l'abaissement, à compter du 1 juillet prochain, de la vitesse maximale autorisée de 90 kilomètres par heure à 80 kilomètres par heure sur les routes à double sens sans séparateur central. Cette décision est loin d'être anodine et concernera, dans la pratique, une part significative du réseau routier secondaire ! Cette mesure a suscité de nombreuses oppositions et critiques. Beaucoup s'interrogent sur son utilité et sur sa proportionnalité. Les incompréhensions parmi la population sont d'autant plus vives que le Gouvernement n'a pas procédé à une concertation préalable suffisante ni fourni d'éléments de nature à étayer sa décision. Selon une étude récente réalisée par l'assureur Axa Prévention, 76 % des Français y seraient ainsi opposés. Or nous savons que l'efficacité d'une mesure repose en partie sur sa compréhension et sur son acceptabilité par la population. Cela est d'autant plus vrai en matière de sécurité routière, domaine dans lequel le comportement des conducteurs joue un rôle majeur. Qui plus est, dans un contexte où la fracture territoriale et le sentiment d'éloignement, déjà éprouvés par beaucoup de nos concitoyens, risquent de s'en trouver exacerbés. Je rappelle, en outre, qu'il est nécessaire d'aborder l'enjeu de la sécurité routière de manière globale, en incluant notamment la question des moyens accordés aux collectivités pour l'entretien et la réfection des routes, ou encore la prévention des conduites à risque telles que l'absorption d'alcool, de stupéfiants ou la prise de certains médicaments.

chargé de conduire ses travaux dans des délais contraints, liés au souhait de rendre des conclusions en temps utile, c'est-à-dire avant la publication du décret de mise en oeuvre de la réduction de vitesse à 80 kilomètres par heure. Nous nous sommes ainsi Nous nous sommes ainsi efforcés d'évaluer, sans, l'utilité et l'efficacité de cette mesure en organisant une série d'auditions, afin d'entendre l'ensemble des parties prenantes : principaux acteurs de la sécurité routière, représentants d'élus locaux, usagers de la route quarante-sept personnes ont été entendues, à l'occasion de dix-sept auditions et tables rondes. Nous avons, en parallèle, décidé d'ouvrir sur le site du Sénat un espace participatif, afin d'associer à cette réflexion l'ensemble de la société civile. Le succès de cette plateforme est sans précédent : en quelques semaines, plus de 23 000 contributions de citoyens ont pu être collectées ! Dans l'ensemble, les témoignages recueillis font état d'un rejet assez large de la mesure au sein de la société civile. S'il est bien sûr difficile de généraliser ces conclusions, nous pouvons, en tout état de cause, y voir le signe d'une très forte mobilisation. Les deux commissions ont adopté à l'unanimité le rapport que nous leur avons soumis le 18 avril dernier. Mes deux collègues vous présenteront de manière plus précise les résultats de nos travaux, ainsi que nos propositions. Je souhaite, à cet égard, rappeler qu'un consensus s'est très naturellement dégagé sur les conclusions de ce rapport. Mes chers collègues, la réduction de la mortalité sur les routes doit, plus que jamais, être placée au rang de priorité. Mais il est de notre devoir de parlementaires de nous assurer que les mesures mises en oeuvre par le Gouvernement sont pertinentes et proportionnées au regard de l'objectif poursuivi. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, permettez-moi de commencer mes deux collègues qui viennent de s'exprimer. Ensemble, nous avons formé un trio qui, je le pense, a travaillé tout à fait honnêtement. Je tiens également à remercier les administrateurs qui nous ont accompagnés tout au long de ces quarante-sept auditions et qui ont rédigé le rapport à votre disposition pour un coût de 3,50 euros, mais qui sera donné gracieusement ! Le 14 juin prochain, les trois rapporteurs du groupe de travail sur la sécurité routière iront défendre leurs travaux et leurs recommandations auprès du Premier ministre Édouard Philippe. Je m'y rendrai avec la ferme volonté de le convaincre de changer ses positions. Il est bien évident que nous partageons les mêmes objectifs : comme mes collègues l'ont dit, chaque mort, chaque blessé est de toute façon un mort ou un blessé de trop. Le débat n'est pas là : il porte sur les moyens et les modalités de mise en oeuvre.

Paradoxe, d'abord, au regard du discours général du Gouvernement vantant les mérites de la concertation et le respect des spécificités des territoires. Ainsi, dans le cadre du nouveau pacte ferroviaire, le rôle des régions est considérablement renforcé, car, nous dit-on, elles connaissent les besoins et les contraintes de leurs territoires. Pourquoi la sécurité routière devrait-elle faire exception ? Sur les limitations de vitesse, notre position n'est pas dogmatique. Pourquoi pas 80 kilomètres par heure là où cela se justifie ? Mais laissons plutôt les départements, gestionnaires des voiries, moduler la vitesse en fonction de critères objectifs

Paradoxe, enfin, d'un Premier ministre qui campe sur des positions fondées sur une étude controversée, et qui ne parvient pas à créer l'unanimité au sein même de son gouvernement.

Avant de conclure, mes chers collègues, et pour être absolument certaine que toutes les conditions seront réunies pour convaincre le Premier ministre, je souhaite lancer deux appels solennels. Le premier s'adresse aux présidents des conseils départementaux.

Le second s'adresse au ministère de l'intérieur. Je sais combien ses effectifs sont mobilisés au service de la République. Pourtant, les résultats d'une politique générale de sécurité routière ne se feront réellement sentir que par une multiplication des contrôles. difficile, pour nos concitoyens, d'accepter des mesures de limitation de vitesse quand ils savent, par ailleurs, que 600 000 automobilistes circulent sans permis ou que les rodéos nocturnes se poursuivent en toute impunité. J'ai la certitude que la vision de notre groupe de travail est la bonne. Encore une fois, nous poursuivons les mêmes objectifs ; seule la mise en oeuvre diffère : nous faisons confiance aux gestionnaires de voirie et au terrain.

une mesure ne se doit pas d'être populaire pour démontrer son efficacité. Mais si nous avons la possibilité de la rendre moins impopulaire sans la rendre inefficace, pourquoi nous en priver ? Madame la ministre, je compte sur vous pour faire entendre raison à M. le Premier ministre. La parole

À la suite du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier dernier, le Gouvernement, par la voix du Premier ministre, a décidé avec ténacité qu'à compter du 1 juillet prochain la vitesse maximale autorisée sur les routes à double sens sans séparateur central serait réduite de 90 kilomètres

« n'avait pas pour but de faire diminuer le nombre de morts ». Heureusement, car ses résultats sont extrêmement mauvais, et ce malgré la réalisation d'importants travaux de sécurité de voirie avant l'expérimentation. Cette mesure n'est justifiée que par un chiffre hypothétique- 400 morts pourraient être évitées - tiré de l'idée selon laquelle une diminution de 1 % de la vitesse entraînerait une baisse de 4 % des accidents mortels.

En l'absence d'éléments de nature à justifier cette décision très contestée par la population, par de nombreux parlementaires de la majorité présidentielle, par les forces de l'ordre dans leur majorité, le Sénat a mis en place un groupe de travail conjoint afin d'évaluer, sans, l'utilité et l'efficacité de cette mesure.

Le ministre de l'intérieur lui-même doute de l'efficacité d'une généralisation de cette mesure. Il a dit « joker », et c'est vous, madame la ministre, qu'il envoie au charbon aujourd'hui

Sur la route, le risque zéro ne peut exister. Nous vous demandons donc, madame la ministre, de prendre en compte les territoires pour lesquels la route est le seul moyen de se déplacer. La politique du tout radar ne marche plus depuis qu'on privilégie le désendettement de l'État plutôt que la sécurité. Notre collègue Vincent Delahaye l'a démontré : la politique d'implantation des radars favorise la rentabilité au détriment

Les dotations versées par l'État aux départements pour l'entretien des routes ne cessent de diminuer, alors même que le produit des radars n'a jamais été aussi élevé. Dans mon département, la Vienne, les dotations ont baissé de 27 % entre 2015 et 2017.

de promouvoir des comportements raisonnables et responsables sur la route, pour toujours plus de sécurité. Quant au choix des routes qui feront l'objet d'une réduction de la vitesse, faisons confiance aux présidents de département ! Madame la ministre, je vous connais, vous êtes convaincante.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, près de 3 700 personnes ont perdu la vie sur les routes de France en 2017, les accidents corporels ont augmenté de plus de 2 %, et le nombre de personnes blessées de 1,3 %, soit près de 74 000 personnes, pour 59 000 accidents ; la situation de la sécurité routière en France est donc préoccupante. son plus bas niveau en 2013, la mortalité routière a connu trois années de hausse consécutives. Pour répondre à cette évolution inquiétante, le Gouvernement a décidé d'abaisser à 80 kilomètres par heure la limitation de vitesse sur les routes nationales à compter du 1 juillet.

Toutefois, le Premier ministre a confirmé l'entrée en vigueur de cette mesure à partir de l'été prochain. La véritable question est donc désormais celle de sa mise en oeuvre concrète et opérationnelle. Le coût de l'installation de la nouvelle signalisation est estimé entre 5 et 10 millions d'euros. Il a été annoncé que ce coût serait entièrement pris en charge par l'État. Par ailleurs, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière et les observatoires départementaux

En tant qu'élue d'un département rural et très enclavé, je suis cette mesure avec une attention particulière. En effet, la plupart des routes concernées se trouvent dans ces territoires où les transports en commun sont peu, voire très peu développés, où certaines petites lignes de chemin de fer pourraient être menacées, et où le véhicule personnel est indispensable pour pouvoir se déplacer. Si l'on ne peut que souscrire à la volonté de lutter sans relâche contre la violence et la mortalité routières, il existe de vraies interrogations et, localement, de fortes,

Malgré le bien-fondé de l'objectif final, il faut convenir que cette limitation contribuera, malheureusement, à aggraver l'enclavement déjà excessif de nos territoires. Cibler l'application de cette mesure m'apparaît donc essentiel. Que les décisions soient prises au plus près du terrain ! De plus, des mesures énergiques doivent être prises afin de modifier durablement les comportements dangereux : il faut interdire le téléphone et les écrans, et assurer le respect des limitations de vitesse. Des investissements doivent également être réalisés afin d'améliorer l'état des routes. La France bénéficie d'infrastructures de transport d'une grande qualité, mais ce réseau est aujourd'hui trop peu entretenu. En outre, du fait de la départementalisation des routes et du manque de compensation financière de l'État, les disparités territoriales ont tendance à s'accroître. La forte baisse des financements à destination des collectivités locales, notamment en raison de la décentralisation du stationnement payant, n'est pas de nature à améliorer la situation. La position du Sénat sur ce point me paraît raisonnable et ses propositions mériteraient d'être expérimentées. Dans tous les cas, la France doit pouvoir trouver les moyens d'améliorer réellement la sécurité routière.

On voit bien que la vitesse n'explique pas tout. Les efforts en matière d'éducation doivent être poursuivis et accentués. Le rapport de Jean-Marc Gabouty sur le programme « Sécurité et éducation routières » de la loi de finances pour 2018 a salué une amélioration de la sincérité budgétaire pour les dépenses de communication les frais d'étude et d'expertise. La réforme du permis de conduire, engagée en 2014 et 2015, semble également porter ses fruits. On peut espérer que, grâce à elle, on verra de moins en moins de jeunes conduire sans permis. Le délai moyen d'attente pour le passage de l'examen du permis de conduire poursuit sa baisse.

Cette réforme semble obtenir des résultats positifs, puisque le délai moyen entre deux présentations à l'examen du permis B est passé de 90 jours en 2014 à 57 jours en 2017. L'objectif d'une attente moyenne de 45 jours, inscrit inscrit au projet annuel de performance de 2017, n'apparaît donc plus hors d'atteinte. Parallèlement, la durée de validité de l'examen du code est passée de trois à cinq ans. Les conditions de distance et de durée minimale pour la conduite accompagnée ont été supprimées, et les recrutements d'inspecteurs du permis de conduire ont été encouragés. En revanche, le coût de la formation et des épreuves pour les usagers continue de poser problème. Selon le rapport remis en 2014 par Mme Florence Gilbert, ce coût s'établit en moyenne à 1 600 euros, ce qui reste un montant très élevé. En sont responsables des frais administratifs encore trop importants et un coût horaire de la leçon de conduite très élevé. Afin de remédier réellement à ces difficultés, la solution ne serait-elle pas d'améliorer la concurrence entre les auto-écoles ou, en cas de défaillance du marché, de nationaliser l'ensemble de la formation, voire d'en faire une matière scolaire ? Je vous remercie, madame la ministre, de répondre à ces différentes interrogations.

année, 3 500 tués et- on a oublié de le rappeler ce soir -75 000 blessés, dont 28 000 grièvement. Ce sont autant de nos concitoyens qui, chaque année, voient leurs vies bouleversées, ainsi que les membres de leurs familles. Tous, nous refusons de nous satisfaire de cet état de fait, nous refusons cette fatalité. Il fallait donc une nouvelle impulsion.

à 80 kilomètres par heure sur les routes secondaires à double sens sans séparateur central, sur lesquelles 55 % des drames se produisent.

le soin de décider de cet abaissement sur les routes les plus accidentogènes. Cette question a été posée de manière réitérée. Gagnerait-on en visibilité ? Je n'en ai pas été convaincu ce soir.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, je tiens d'abord à remercier mes collègues rapporteurs pour leur travail. Depuis le début du siècle, les efforts se multiplient pour améliorer la sécurité sur nos routes et, ainsi, épargner des vies humaines. Dans un contexte de recrudescence du nombre de tués sur nos routes, le Gouvernement a proposé un nouveau plan de renforcement de la sécurité routière.

Cette mesure, décidée hâtivement et sans concertation avec les territoires, aura, de mon point de vue, surtout servi à créer un écran de fumée pour occulter la désastreuse politique gouvernementale. La réduction de la vitesse permettra certainement de sauver des vies et aura un aspect pédagogique, mais une démarche plus ciblée en concertation avec les acteurs locaux aurait été préférable et plus efficace.

effet- ce sera le coeur de mon intervention -, je déplore que ni la mission sénatoriale ni le plan gouvernemental n'aient sérieusement pris en compte la sécurité, sur nos routes, de tous les usagers, et plus particulièrement des cyclistes. Pour être précis, la seule mesure du plan gouvernemental qui concerne le vélo n'est qu'une petite généralisation du « savoir rouler », comme si les cyclistes, usagers de la route les plus fragiles, étaient responsables de leurs propres accidents mortels J'entends déjà des murmures me suggérer que cet enjeu est marginal, anodin, voire hors sujet. Détrompez-vous, mes chers collègues : l'usage de la route change ! L'usage du vélo est en constante progression pour des raisons économiques, écologiques et sanitaires. De plus en plus de nos concitoyens remplacent la voiture par le vélo pour tout ou partie de leurs déplacements. Le déploiement du vélo électrique décuple ce phénomène. En effet, il permet d'effectuer sans trop d'efforts des trajets de plusieurs dizaines de kilomètres, quelle que soit la topographie. Même en zone rurale, même dans les montagnes du Trièves d'où je viens, faire à vélo le trajet entre domicile et travail n'est plus réservé aux athlètes. Pourtant, nos routes ne sont pas du tout adaptées à la pratique du vélo et demeurent dangereuses pour les cyclistes. Rappelons que les deux tiers des cyclistes tués sur la route le sont en dehors des agglomérations.

Je déplore que cette loi soit si souvent contournée par les collectivités ou appliquée dans sa version minimale, en dessinant une simple bande cyclable sur la droite de la chaussée. Notons qu'une bande cyclable sans séparateur est contre-productive, car elle élargit la chaussée et invite l'automobiliste à rouler plus vite au détriment de la sécurité des cyclistes qui l'empruntent. Vingt-deux ans après, tant pour des raisons écologiques que pour des raisons de sécurité, il faut renforcer la rédaction de la loi LAURE et imposer des aménagements cyclables dignes de ce nom,

Il est dommageable de dissocier les problématiques de sécurité routière de celles de qualité des infrastructures. Il ne fait pas de doute qu'une chaussée dégradée est un facteur d'insécurité, tout comme l'est une voie ferrée endommagée. Le Gouvernement nous renverra à sa future loi de programmation des infrastructures, limitant la portée de ce nouveau plan. La question financière est ici primordiale, car l'entretien de la voirie coûte cher et demeure à la charge des seules collectivités. Celles-ci, déjà exsangues, ne sont pas toujours en mesure de réaliser d'indispensables réfections. Il est donc nécessaire de les épauler. Cela passe par la mise à contribution-

Pour revenir à des sujets relevant du ministère de l'intérieur et ne demandant pas de lourds investissements, le Gouvernement peut tout de même prendre des mesures pour améliorer la sécurité des cyclistes. Par exemple, nous pourrions imposer aux constructeurs d'abonder un fonds de formation continue des conducteurs ayant obtenu leur permis il y a plus de cinq ans.

Enfin, il faut intensifier la verbalisation des infractions de non-respect des aménagements cyclistes, qui peuvent avoir une conséquence importante en matière de sécurité. Madame la ministre, mes chers collègues, le vélo ne peut plus rester le parent pauvre des politiques de sécurité routière. C'est pourquoi je vous invite à avancer en ce sens. La

La sécurité routière est un impératif, il n'y a pas de débat là-dessus. Il est toutefois possible de réduire l'insécurité routière sans porter atteinte au quotidien des habitants et en écoutant les représentants de la Nation et les citoyens, qui sont les premiers concernés Réduire la vitesse maximale autorisée à 80 kilomètres par heure sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central, la mesure est justifiée. Reste que votre manière de faire et de mettre en place cette mesure est dénuée de pragmatisme : une fois de plus, vous avez préféré agir de manière soudaine et imposer. et imposer. Au lieu d'écouter et d'adapter cette mesure aux routes accidentogènes, vous persistez à tout imposer d'en haut, et sur tout le réseau routier départemental. Pourtant, nombreux sont ceux qui se sont exprimés, au sein de la société civile et parmi les élus locaux, contre la généralisation d'une telle mesure, dont l'utilité et l'efficacité sont, pour beaucoup, loin d'être certaines. L'Association des maires de France et l'Assemblée des départements de France, qui

d'information du Sénat sur la sécurité routière n'est pas seulement un travail d'élus, qui sont certes représentants de la Nation. Les sénateurs ont aussi mis en place un espace participatif afin d'associer à leur réflexion l'ensemble de la société civile : des dizaines de milliers de contributions ont été reçues.

Une telle mesure de réduction généralisée, qui touchera sans discernement la majorité des routes nationales et départementales hors agglomération, est ainsi très mal vécue sur de nombreux territoires enclavés, où la route est une infrastructure de mobilité incontournable. Cette mesure est perçue comme d'autant plus injuste que les services de l'État ont parfois refusé, dans ces territoires, d'aménager les routes nationales afin de les transformer en routes à deux fois deux voies. vous agissez comme si vous pensiez que les territoires ne pouvaient pas et ne savaient pas gérer. Pourtant, dans ce domaine, la pertinence de l'action n'est pas seulement centralisée, elle est aussi territoriale et départementale. Quelle contradiction, monsieur de Belenet ! Vous acceptez que les maires décident pour les zones urbaines, mais n'acceptez pas que les présidents de conseil départemental décident pour les zones rurales. La base de la circulation routière, donc de la sécurité routière, ce sont assurément les infrastructures et leur état. Si une route est en mauvais état, les bases manquent pour une conduite en toute sécurité. Notre patrimoine routier est dégradé, cela a été répété à cette tribune

plus de 85 % de chaussées étaient dans un état correct entre 2010 et 2012, ce chiffre est tombé à 83 % en 2015 », ce qui entraîne « des ralentissements, des restrictions de circulation et des problèmes de sécurité ». je souhaite vous faire part d'un exemple que je connais bien, la RD 2089 entre Clermont-Ferrand et les départements du Cantal et de la Corrèze. Dans les années 2000, on recensait dix à quinze morts par an,

par la construction de créneaux de dépassement, de portions à trois voies, ... Eh oui ! ... de bandes d'arrêt d'urgence et de mini-échangeurs aux croisements dangereux, ainsi que des opérations de sécurité, et toujours à 90 kilomètres ! Madame la ministre, donnez-nous les moyens d'améliorer ce réseau routier. Par ailleurs, vous agissez comme si vous ne voyiez pas que les technologies automobiles avaient évolué et allaient encore considérablement le faire à l'avenir.

Il serait primordial de les mettre en place désormais et non de se focaliser sur une seule proposition qui suscite une opposition quasi unanime et dont vous ne saurez jamais si elle a permis la diminution du nombre de tués sur les routes départementales. En outre, le groupe de travail sénatorial considère que le surplus financier qui serait issu de la réduction de la vitesse maximale autorisée à 80 kilomètres par heure sur certaines routes devrait être alloué au financement de mesures de prévention, par exemple de sensibilisation. La proposition du Sénat est raisonnable, intelligente et acceptable. Après les zones 30, laissez les acteurs du terrain mettre en place les zones 80, afin que la réduction de la vitesse obtienne des résultats efficients et certains pour la sécurité routière et la sécurité de chacun. chacun. Madame la ministre, n'allez pas à 100 à l'heure : écoutez les acteurs du territoire et les citoyens ! C'est maintenant que vous avez rendez-vous avec eux et non dans deux ans. La parole est à M. Olivier Cigolotti. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, comme nous le savons tous, depuis quarante ans, les efforts conjugués réalisés en matière de sécurité routière ont permis une baisse quasi continue des accidents de la route, du nombre de blessés et de morts, et ce en dépit d'une augmentation considérable du nombre de véhicules et des kilomètres parcourus. En effet, dans les années 1970, nous recensions environ 17 000 morts sur les routes pour un parc automobile d'environ 13 millions de véhicules particuliers. En 2017, pour 32 millions de véhicules particuliers en circulation, c'est un peu moins de 4 000 décès, soit quatre fois moins. Certes, c'est encore trop. Cette nette diminution tient autant, voire plus, à des éléments techniques, culturels et psychologiques qu'à la seule efficacité de la répression et de la peur du gendarme, même si cette dernière a évidemment joué un rôle certain. Un ensemble de facteurs ont réduit le nombre d'accidents et leurs conséquences. Je pense à l'amélioration continue de la tenue de route des véhicules, de la résistance aux chocs, du freinage, des pneumatiques ; je pense encore au port de la ceinture de sécurité,

Ce constat nous oblige à considérer les enjeux de sécurité routière comme une question large et multifactorielle, qui ne doit surtout pas se limiter à la seule donnée de la vitesse autorisée sur les routes. Je tiens à saluer le travail nuancé et objectif réalisé par nos trois rapporteurs, Michèle Vullien, Jean-Luc Fichet et Michel Raison, sur les mesures destinées à renforcer la sécurité routière. Cet excellent rapport d'information a notamment pu mettre l'accent sur deux points essentiels d'une part, la nécessité de revoir la méthode retenue par le Gouvernement ; d'autre part, le manque de concertation ayant présidé à la décision de limiter à 80 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée sur les 400 000 kilomètres de routes secondaires à double sens sans séparateur central, qui devrait entrer en vigueur à partir du 1 juillet prochain. Selon certaines sources, 76 % des Français y sont opposés. Si la diminution du nombre de victimes d'accidents de la route est un objectif que l'on ne peut que partager, cette décision de réduire la vitesse, dont la pertinence reste à démontrer, est d'autant plus mal vécue qu'elle a été prise sans concertation, ... Exactement ! C'est bizarre ! ... sans que les bénéfices en termes de sécurité routière aient fait l'objet d'évaluations sérieuses et, de toute évidence, en sous-estimant les conséquences en matière d'aménagement du territoire. Cette limitation de vitesse suscite donc la colère et l'incompréhension d'un grand nombre d'usagers de la route et d'élus, particulièrement des habitants des zones rurales qui la vivent comme une

éloignées des autoroutes et des grandes métropoles et souvent mal desservies par le réseau ferroviaire, et les zones urbaines ou périurbaines. Il me semble évident que les difficultés de déplacement dans les territoires ruraux ne sont aucunement prises en compte dans cet arbitrage. Je pense par exemple aux zones de montagne, dont le réseau routier sera largement concerné par cette réduction de vitesse, ou encore aux départements qui n'ont pas la chance de bénéficier d'infrastructures routières modernes à deux fois deux voies, qui ne disposent pas de transports collectifs routiers ou ferroviaires et où la seule solution consiste à utiliser un véhicule personnel pour se déplacer. Certains arguments, tels qu'une réduction de la pollution, sont également avancés pour justifier la nécessité de réduire la vitesse. Cependant, les études menées par des organismes de surveillance de la qualité de l'air montrent que passer d'une vitesse de 90 kilomètres par heure entraîne un rejet plus important de composés organiques volatils et n'a qu'un impact minime sur les émissions d'oxyde d'azote. Sans compter que, plus l'on passe de temps sur la route, plus l'on pollue. L'axe central avancé par la Sécurité routière pour justifier cette mesure est celui de la vitesse, celle-ci étant présentée comme la première cause de mortalité. La détermination de la causalité des accidents corporels n'est pourtant pas chose aisée. Certains facteurs accidentogènes, comme la vitesse, sont souvent identifiés par défaut, ce qui nuit nécessairement à la fiabilité des données produites. Les accidents trouvent souvent leurs origines dans une combinaison multifactorielle- alcool, stupéfiants, téléphone, endormissement sans oublier les conduites addictives. À cela s'ajoute le non-respect des autres règles de circulation, généralement à l'origine d'une part significative des accidents. Notons, de plus, que le facteur lié à l'infrastructure est présent dans 40 % des accidents mortels. Isoler le facteur vitesse pour réduire la mortalité sur les routes n'a donc vraiment pas de sens. Force est de constater que cela pourrait même augmenter les risques pour les conducteurs, puisque les voitures et les motos rouleront à la même vitesse que les camions, ce qui multipliera le risque de dépassement dangereux. J'en viens aux radars. La France compte 4 600 radars avec des modèles de plus en plus perfectionnés. Oui ! Or, nous le savons tous, une baisse de la limitation de vitesse entraînera inéluctablement un doublement, voire un triplement des excès de vitesse. Un rapport de la Cour des comptes fait le point sur ces flashs, qui rapportent chaque année davantage à l'État : 1 milliard d'euros en 2017, soit 10 % de plus que l'année précédente. Cette recette permet de renforcer la sécurité routière et, certes, de financer une partie des préjudices. La Cour des comptes s'interroge toutefois sur l'utilisation des amendes, qui participent davantage au remboursement de la dette qu'au financement de la sécurité routière. Il ne faudrait donc pas que cette limitation de vitesse ait pour unique objectif de remplir les caisses de l'État. Eh si ! Bravo ! Madame la ministre, alors que le Gouvernement cherche à redonner confiance à l'échelon local en prenant en compte un certain nombre de spécificités et à décliner à l'échelon départemental la police de sécurité du quotidien- la PSQ, dont tout le monde entend parler actuellement le même ministère, le vôtre, agit aujourd'hui avec incohérence en souhaitant généraliser une réduction de vitesse, qui mérite pourtant, d'une part, d'être ciblée sur les routes les plus accidentogènes à travers des décisions décentralisées, d'autre part, d'être adaptée en fonction des réalités des territoires, lesquels devraient être associés à cette prise de décision, en concertation avec l'ensemble des acteurs, afin d'en favoriser l'acceptation. Madame la ministre, vous connaissez le bon sens du Sénat. Nous comptons sur vous pour relayer l'excellent travail de la Haute Assemblée auprès de M. le Premier ministre. C'est déjà fait ! Cigolotti

J'entends les critiques sur le déficit de concertation et sur le sentiment de mépris des territoires et je dois dire qu'elles ne sont pas sans fondement. Il faut toutefois constater que, à chaque mesure prise par les pouvoirs publics pour réduire la mortalité sur les routes, depuis l'obligation du port de la ceinture de sécurité en 1973 à la mise en place des radars automatiques en 2003, des voix se sont élevées pour critiquer en usant de tous les arguments possibles.

J'entends la recommandation faite par nos collègues rapporteurs visant à décentraliser et à adapter la mesure en fonction des territoires, mais je ne suis pas certain qu'elle qu'elle soit efficace. Si je peux en partager l'idée et le principe, je pense que son application risque d'être contre-productive. Il est plus simple pour les usagers de la route, dans quelque domaine que ce soit, et plus efficace pour l'objectif que nous souhaitons atteindre de bénéficier d'une règle générale et de quelques exceptions : une règle simple, c'est un message fort, c'est un message compris. Or la décentralisation de cette règle ne risquerait-elle pas d'entraîner une très grande diversité de limitations, renforçant l'imprévisibilité pour les usagers ? Nous ne pouvons pas faire abstraction de cette interrogation.

Il faut davantage lutter contre l'utilisation du téléphone au volant, contre la consommation d'alcool et de stupéfiants. Ces combats doivent être livrés de façon plus active.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, j'évoquerai deux sujets concrets, qui ont un impact direct sur la sécurité routière et, plus généralement, sur la sécurité de nos concitoyens

Entre 2015 et 2016, les recettes liées aux radars ont progressé de plus de 13 millions d'euros, pour atteindre les 920 millions d'euros. Dans le même temps, la mortalité routière n'a cessé de croître, et ce pour la troisième année consécutive, portant à près de 3 500 le nombre de tués pour la seule année 2016. La vitesse n'en est pas la seule et principale cause, loin de là. Les Français en ont assez d'être pris pour des vaches à lait

J'ajoute que cette mesure sortie du chapeau a été prise sans concertation : ni les élus locaux ni les préfets n'ont été consultés. Bien pis, elle ne repose que sur des données très contestables. d'État, ministre de l'intérieur, va-t-il sérieusement remplacer les quelque 20 000 panneaux 90 ou 90 barré ? Allez-vous sérieusement engager la France dans une telle dépense ? Le Premier ministre a annoncé que, au 1 juillet 2020, le Gouvernement tirerait les conséquences de cette mesure. Quelle absurdité de prendre le risque de devoir changer de nouveau tous les panneaux dans deux ans ! Je crois que, au fond de lui-même, le ministre de l'intérieur n'est pas convaincu par cette mesure stupide- peut-être ne l'êtes-vous pas vous-même, madame le secrétaire d'État parce que l'expérimentation n'a pas fait ses preuves, parce qu'elle est coûteuse, parce qu'elle est pénalisante pour nos territoires,

C'est vrai qu'on aurait pu regarder les tranches les plus accidentogènes ». Eh bien, je suis d'accord avec M. le ministre d'État : nous devons procéder par sectorisation. Laissons aux départements le soin de déterminer les portions où la vitesse doit être baissée à 80 kilomètres par heure et celles où la vitesse doit demeurer à 90 kilomètres Emmanuel Macron lui-même disait, lorsqu'il était encore candidat : « En France, les vitesses sont impaires : 30, 50, 70, 90, 110, 130. Cela participe de leur lisibilité. Je suis naturellement favorable, dès lors que les conditions de danger l'imposent, à abaisser la vitesse à 70, » ... Évidemment ! ... « mais abaisser en section courante la vitesse à 80 interrogerait l'ensemble de l'édifice. » Voilà ! Madame le secrétaire d'État, trois fois, mais je le répète volontairement ! ... vous qui avez été longtemps une élue locale, ayez la volonté de dire au Président le mal que les territoires pensent de cette décision. Il décide tout seul ! L'alcoolisme, les fautes de comportement sont plus mortels que la vitesse. Si les Français se désintéressent de plus en plus de la politique, c'est à cause du double discours permanent que leur servent une poignée de responsables publics. Je souhaite maintenant évoquer avec vous un second sujet, qui est lié à la sécurité générale, donc à la sécurité routière. La loi du 3 juin 2016 et son décret du 23 décembre de la même année ont autorisé, à titre expérimental, pendant deux ans, l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions, y compris sur les routes. Tous les élus locaux et tous les policiers municipaux que je rencontre sont pleinement satisfaits de cette disposition. Le port d'une caméra individuelle est d'ailleurs assez répandu. Il est autorisé à la fois pour les policiers, les gendarmes, même les agents de la SNCF et de la RATP, et certainement, très bientôt, les pompiers. De l'avis unanime des acteurs de terrain, cette mesure ne présente que des avantages. Elle est d'abord une garantie pour la procédure pénale et les parties concernées. L'encadrement législatif et réglementaire est strict. La preuve collectée aide au constat des infractions et à la poursuite des auteurs. Surtout, elle est une garantie pour nos polices municipales filmer les échanges entre forces de l'ordre et population diminue les tensions et les incivilités. C'est aussi une protection contre les mises en cause. Enfin, c'est un témoin contre les agressions et les outrages subis par nos agents. Pourtant, madame la ministre, malgré toutes les garanties que présente le port d'une caméra dite « piétonne », rien n'a été prévu par votre gouvernement pour pérenniser ce dispositif. Concrètement, cela veut dire que, depuis le 3 juin de cette année, les policiers municipaux ont dû renoncer à utiliser leurs caméras, lesquelles ont été financées- ce sont des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros -par des subventions d'État.

c'est un manque de considération pour les parlementaires, mais c'est aussi une mauvaise manière faite aux Français automobilistes à qui l'on impose un oukase, par définition à contre-pied d'une démocratie de proximité. La parole est

Cette énergie acquise doit être dissipée pour que le véhicule s'arrête. En d'autres termes, celui-ci ne s'arrêtera que lorsque toute l'énergie sera dissipée et transformée. Si le freinage est impossible ou insuffisant, l'énergie se dissipera par destruction, ce qui peut entraîner des blessures, voire le décès des passagers.

et pour que l'inventivité et la créativité dont nous sommes capables soient à l'origine de mesures plus adaptées. Si la vitesse aggrave incontestablement les accidents, il faut aussi s'interroger sur les relations causales que sont le non-respect du code de la route, le degré d'alcoolémie, l'usage des stupéfiants, des médicaments, du téléphone, la fatigue, la somnolence, le rôle des camions ou encore le mauvais entretien des routes.

durable oblige, il y aura davantage de piétons et cyclistes, il faudrait y réfléchir sérieusement. La mortalité routière connaît en France une stagnation depuis quelques années. La sécurité routière doit s'élever au haut rang des politiques publiques prioritaires.

Or l'expérimentation n'a pas mesuré l'évolution de l'accidentalité, n'a pas étudié en parallèle des tronçons sans limitation pour servir de témoins. En outre, elle s'est limitée à seulement quatre semaines. Je ne contesterais pas non plus cette réforme, si elle n'était pas à double tranchant pour nombre de nos territoires. Cette mesure, madame la ministre, devrait bien entendu s'appliquer dans le cadre de la décentralisation, donc au cas par cas. La loi de décentralisation du 13 août 2004 a abouti au transfert d'une certaine partie du réseau routier national aux départements. Aujourd'hui, vous nous annoncez une mesure qui aurait dû être, si ce n'est laissée à la discrétion et à l'appréciation des départements, au moins concertée avec ces derniers. Je plaide donc, pour reprendre les mots du rapport d'information présenté par nos collègues, pour la mise en place de « conférences départementales de la sécurité routière », qui seraient coprésidées par les présidents de conseil départemental et les préfets et « dont le rôle serait d'identifier les routes ou les tronçons de route accidentogènes

les accidents se concentrent à 65 % sur le réseau principal, le réseau secondaire ne représentant que 25 % des accidents. Notre département se caractérise par un niveau d'investissement dans la voirie supérieur à la moyenne des collectivités de sa strate.

essentiel. La sécurité routière nous concerne tous et mérite une politique publique sérieuse, adaptée et efficace. À titre personnel, je le mesure d'autant plus que le nombre d'accidents corporels et de morts sur les routes dans mon département de Maine-et-Loire est significativement supérieur à la moyenne nationale depuis plusieurs années. La sécurité routière est l'affaire de tous, tant des élus que des associations qui oeuvrent au quotidien pour la prévention. Le travail des sénateurs sur ce sujet est bien loin d'être une simple posture politique. Il relève au contraire de la recherche d'efficacité et de résultats. À cet égard, je remercie les rapporteurs Michel Raison, Michèle Vullien et Jean-Luc Fichet de leur travail. Je salue notamment l'investissement de mon collègue Michel Raison,

Tout cela n'est en réalité pas très sérieux. Nous attendons une politique bien plus ambitieuse. Il conviendrait notamment d'activer d'autres leviers comme l'éducation et la prévention. Cette réduction généralisée, qui ne prend en compte ni l'état des routes ni leur tracé, est aberrante pour bon nombre de nos concitoyens, cela a été rappelé. En tant qu'élus En tant qu'élus de terrain, nous le ressentons dans nos départements : l'exaspération est réelle et ne cesse de croître. L'impression, en toile de fond, est qu'il s'agit là d'une vision purement parisienne, déconnectée des réalités et sans véritable fondement. Or, vous le savez comme nous, lorsqu'une mesure n'est pas adaptée et n'est pas comprise, elle n'est pas respectée. La véritable question qu'il convient de se poser est celle de l'adéquation entre une limitation de vitesse et la route à laquelle elle s'applique.

! Imposer une même limitation sur toutes les routes c'est nier la capacité d'appréciation des autorités locales. Madame la ministre, pourquoi vous entêtez-vous à ignorer l'avis des acteurs de terrain ? Pourquoi avez-vous tant de mal à faire confiance aux élus ? Il est encore temps d'aménager le dispositif et de mettre en place une réglementation au cas par cas, comme le préconise ce rapport et comme le souhaitent les présidents de département. Les automobilistes français méritent une politique de sécurité routière réfléchie, ambitieuse et efficace. J'espère que le Gouvernement entendra l'appel des élus locaux

sous la présidence du Premier ministre, par le Conseil interministériel de la sécurité routière le 9 janvier 2018.

la réduction de la vitesse maximale autorisée, son effet sur la baisse des vitesses pratiquées et, de fait, sur la mortalité. Je relève en effet que les rapporteurs proposent non pas de rejeter en bloc la mesure, mais de ne l'appliquer que sur les routes ou les tronçons de route les plus accidentogènes, en fonction de leurs caractéristiques et de leur environnement.

de loi sur les rodéos, que le Gouvernement soutient, a été déposée par le sénateur de l'Essonne,

L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, l'ONISR, organisme statistique indépendant rattaché au délégué interministériel à la sécurité routière, l'a démontré dans un rapport publié le 17 avril dernier, peu avant le dépôt de votre rapport. Il est intéressant de disposer de ces rapports sur l'état de la situation.

Aucun département n'échappe à cette règle

Si l'on ajoute à ces 10 % le réseau un peu moins important, qui est en moyenne de 10 %, on constate que, sur 20 % du réseau, on déplore 55 % des tués.

le réseau structurant représente 8 % du réseau et 61 % des tués. Si on ajoute le deuxième niveau, sur 18 % des routes du département on dénombre 74 % des tués.

tués. Dans le Finistère, enfin, le premier niveau représente 37 % du réseau, mais concentre 60 % des tués. Ainsi, les réseaux les plus empruntés sont ceux où l'on compte le plus d'accidents parce qu'ils concentrent les risques

En revanche, quand il fait beau, en journée, que la route est sèche, belle et droite, on accélère, on augmente le risque et on y meurt plus souvent, notamment s'il n'y a pas de séparation centrale.

qui connaissent leur réseau. Il n'est donc pas besoin, comme vous le proposez, de différer la mesure et de modifier le réseau auquel elle doit s'appliquer. Ne pas appliquer la mesure à tout ou partie du réseau sur lequel on constate le plus grand nombre de décès serait incompréhensible.

des routes bidirectionnelles sans séparateur central, exception faite des tronçons à quatre voies, ou à trois pour le seul sens du créneau de dépassement où le dépassement peut se faire avec moins de risques.

un dernier point pour finir : certains ont accusé le Gouvernement de vouloir, par cette mesure, gagner de l'argent, combler la dette,

de sécurité du quotidien, vous le savez, tendant à organiser territorialement la sécurité

de son propos. La lutte contre l'insécurité routière est un combat que nous partageons tous dans cet hémicycle, mais c'est un combat qui, pour être efficace, ne peut être mené sans faire oeuvre de pédagogie et sans rechercher un minimum d'adhésion de la part des usagers de la route. Aujourd'hui, force est de constater que les politiques de sécurité routière sont beaucoup trop souvent perçues comme punitives, ce que nous déplorons tous. Pire, beaucoup de Françaises et de Français considèrent que ces politiques ont pour seul objectif de « remplir les caisses de l'État », « de faire du chiffre », disent certains, quand ils ne parlent pas de « racket ». Ce n'est évidemment pas satisfaisant, mais cela illustre bien la défiance à l'égard de la politique de sécurité routière. La décision du Premier ministre- je dis bien du Premier ministre, puisqu'elle ne semble pas faire l'unanimité au sein du Gouvernement -de réduire de manière unilatérale et brutale la vitesse maximale autorisée à 80 kilomètres par heure sur la quasi-totalité des routes secondaires ne fait que renforcer ce sentiment. Cette décision provoque l'incompréhension et le mécontentement de nombreux citoyens et d'élus. Cette incompréhension et ce mécontentement, cette colère même, touchent particulièrement les habitants des territoires ruraux, car ce sont bien eux les plus concernés. Les habitants des grandes villes ou des grandes métropoles disposent en effet de transports en commun pour circuler et, quand bien même ils utilisent leur véhicule, la question de rouler à 90 ou à 80 kilomètres par heure ne se pose pas. En revanche, en milieu rural, vous n'avez pas d'alternative à l'usage de la voiture pour parcourir chaque jour parfois plusieurs dizaines de kilomètres pour aller travailler. Comment s'étonner dès lors que cette mesure soit perçue comme un mauvais coup supplémentaire porté à la ruralité ? Cette mesure est d'autant moins compréhensible qu'elle intervient après la conduite d'une expérimentation dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle est fortement contestée sur le plan scientifique. Le délégué interministériel à la sécurité routière a d'ailleurs été dans l'incapacité d'apporter à nos commissions des éléments tangibles prouvant l'utilité de cette proposition. Le Gouvernement n'y est pas non plus parvenu. Dans ces conditions, pourquoi ne pas avoir commencé par réaliser une véritable expérimentation sur un nombre significatif de tronçons routiers et pendant une période suffisante ? Pourquoi ne pas avoir décidé d'associer le plus largement possible les acteurs concernés à la décision de réduction de la vitesse maximale autorisée, notamment les présidents de département ? À ce problème de méthode s'ajoute un problème lié au caractère uniforme de cette mesure. Une étude publiée par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière le 17 avril dernier, dont vous avez d'ailleurs parlé, madame la ministre, montre que, parmi les routes à double sens sans séparateur central, ce sont les routes nationales et les principales routes départementales drainant le plus fort trafic qui sont responsables du plus grand nombre d'accidents mortels. En approfondissant ce travail, il aurait été possible de dresser une cartographie des routes accidentogènes département par département. Pourquoi, dès lors, vouloir appliquer la réduction de vitesse à l'ensemble des routes bidirectionnelles ? Qui peut prétendre que toutes les routes nécessitent la même limitation de vitesse ? Qui peut affirmer qu'elles présentent toutes la même dangerosité ? C'est pour le moins une vision manichéenne et technocratique. Les propositions formulées par nos rapporteurs, notamment celle de laisser aux présidents de département le soin de fixer la vitesse maximale autorisée en fonction de la dangerosité des routes, me semblent tellement plus logiques et mieux adaptées que ce que le Premier ministre a décidé. Pourquoi refuser d'en tenir compte ? Nous ne pouvons donc que regretter cette décision, madame la ministre, et le fait que le Gouvernement, comme souvent malheureusement, ne fasse aucun cas des travaux menés par le groupe de travail sénatorial. Nos rapporteurs ont formulé une proposition de bon sens qui favoriserait l'acceptabilité de la mesure de réduction de la vitesse maximale autorisée et la rendrait plus efficace. Nous sommes prêts, nous l'avons dit, à soutenir les initiatives du Gouvernement en matière de sécurité routière et sommes majoritairement favorables aux mesures contenues dans le plan visant à renforcer les sanctions contre les auteurs d'infractions graves au code de la route et à sévir davantage contre l'usage du téléphone et l'alcoolémie au volant. En revanche, vous l'avez compris, nous regrettons le caractère général de la réduction de la vitesse à 80 kilomètres par heure, la méthode choisie et l'entêtement du Premier ministre.

Lorsqu'il s'agit de mesures aussi significatives que l'abaissement de la vitesse autorisée sur l'ensemble du réseau, la moindre des choses est de faire preuve de pédagogie et de concertation. Le Gouvernement n'a fait preuve ni de l'une ni de l'autre. Cette mesure ne fera donc que renforcer davantage encore la défiance des Français à l'égard de la politique de sécurité routière et la colère des automobilistes qui vont être verbalisés, particulièrement en milieu rural. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, mes chers collègues, je veux à mon tour saluer et remercier nos rapporteurs qui, en un temps record, ont mené à bien des travaux dont chacun, à cette tribune, a pu saluer la sérénité, l'objectivité, la sagesse, le recul et la hauteur de vue. Madame la ministre, si je partageais vos certitudes, je n'hésiterais pas à soutenir les dispositions que le Premier ministre a arrêtées, mais je ne les partage pas. Le rapport que nos collègues nous ont présenté devrait suffire à convaincre le Gouvernement qu'il a adopté une mesure qui ne produira pas les effets escomptés. La croyance dans l'efficacité de cette mesure me paraît relever d'un acte de foi- j'y suis sensible, bien sûr -plutôt que d'une démonstration. Le rapport d'avril dernier que vous avez cité a parfaitement identifié un certain nombre d'axes sur lesquels les accidents mortels sont nombreux, mais il n'a nullement dit que ces accidents avaient été causés par une vitesse comprise entre 80 et 90 kilomètres

Nous vous rejoignons, bien sûr, pour dire que, sur ces axes, des mesures doivent être prises pour réduire ces accidents. Madame la ministre, vous le savez, j'étais aux côtés de Jacques Chirac quand il a fait de la lutte contre la mortalité routière l'un des grands chantiers de son quinquennat. Je veux vous dire mon engagement total pour cette cause, qui est une grande cause nationale. Nous la partageons tous : il n'y a pas, d'un côté, le Gouvernement qui veut réduire la mortalité routière et, de l'autre, le Sénat

intentions. Le Gouvernement nous dit vouloir s'inscrire, par les mesures nouvelles qu'il propose, dans la continuité de l'action qui a été conduite au début des années 2000. Je ne conteste naturellement ni sa sincérité ni la légitimité de ses intentions, mais il ne suffit pas que les objectifs soient justes pour que les moyens soient bons. Le Gouvernement doit cesser de diaboliser les interrogations et les réserves qui sont exprimées. Elles ne résultent pas d'une résurgence tardive de je ne sais quel poujadisme, mais d'un examen critique, approfondi, documenté, de la pertinence des mesures de limitation de la vitesse normale sur les routes départementales à 80 kilomètres par heure et de l'évaluation de son efficacité. Nous partageons la certitude objective que la vitesse tue. il serait plus exact de dire que c'est l'excès de vitesse par rapport aux limitations actuelles qui tue et non pas le fait que ces limitations seraient insuffisantes. Il n'y a pas de rationalité

les stupéfiants, l'endormissement, l'usage du téléphone portable, les fautes de conduite ... Nos rapporteurs ont réalisé un travail considérable. Ils ont démontré qu'il faut agir sur tous ces facteurs pour être efficace. C'est la proposition qu'ils font avec une mesure

évaluée avant d'être appliquée. La sagesse voudrait que cette proposition soit acceptée par le Gouvernement : c'est une chance que nous lui offrons, une main que nous lui tendons. Notre but ne doit pas être de créer un électrochoc éphémère chez les Français, mais de les faire concourir par adhésion, en obtenant l'évolution de leur comportement au volant, à l'amélioration générale de la sécurité routière.